demande du Gouvernement, l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà près de quatre ans, notre hémicycle avait largement complété la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), afin, notamment, de renforcer le principe de responsabilité élargie des producteurs Nous voici réunis aujourd'hui pour parachever un travail parlementaire au terme duquel nous avons collectivement garanti l'intégrité de ce principe si important pour nos collectivités territoriales et la protection de l'environnement. Ce n'était pas gagné d'avance, car, dans sa version initiale, le texte proposé par l'Assemblée nationale allait à l'encontre de tout ce que nous avions essayé de construire depuis des années en matière d'économie circulaire.

C'était un dangereux précédent susceptible d'affaiblir l'ensemble des REP et, partant, le financement du service public de gestion des déchets. D'autres secteurs auraient, à l'exemple de ce premier régime d'exception, demandé des aménagements et des exonérations pour l'avenir, au détriment des collectivités territoriales et de la protection de l'environnement. Nous ne pouvions pas accepter une telle régression. Nous avons, fort heureusement, parcouru beaucoup de chemin depuis le dépôt du texte à l'Assemblée nationale. Nous le devons au travail engagé dans cet hémicycle. À cet égard, je remercie tout particulièrement les membres de la commission de la culture, en particulier le président Laurent Lafon et notre collègue Michel Laugier leur sens de l'écoute et du dialogue ont grandement contribué à la qualité de nos travaux en première lecture et au caractère équilibré de la solution, exigeante du point de vue environnemental et protectrice de la presse, que nous avons retenue et que la commission mixte paritaire a confortée. Notre priorité était de préserver les filières REP pour protéger le service public de gestion des déchets et nos collectivités territoriales. Cette mission a été accomplie avec le maintien de la presse dans le champ de la REP. Notre seconde priorité était d'aider la presse : c'est aussi chose faite, avec la possibilité, introduite dans le texte sénatorial et conservée par la commission mixte paritaire, de moduler les contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts. le dispositif que nous avions adopté n'a été que légèrement ajusté, afin d'en assurer la sécurité juridique et d'en clarifier la rédaction. Il a ainsi été précisé que le mécanisme adopté ne devra pas conduire à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Pour éviter tout détournement, la rédaction de compromis vise à prévoir, par ailleurs, que les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets ne pourront pas avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. Par cohérence avec la fusion des filières REP, le texte a enfin été modifié pour renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les taux de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion, qui ne pourront, en tout état de cause, pas être inférieurs aux niveaux actuellement prévus par la loi, soit 80 % pour les emballages et 50 % pour les papiers. La balle est maintenant dans le camp du pouvoir réglementaire, qui devra s'assurer du maintien de cet équilibre dans l'application du texte. Notre commission y veillera ! La parole

Après une commission mixte paritaire conclusive, lors de laquelle s'est construit un véritable consensus entre les chambres, nous nous retrouvons aujourd'hui pour soumettre au vote cet accord.

mois de janvier dernier, ce texte prouve encore une fois qu'en faisant confiance au dialogue, il est possible d'aboutir à une rédaction qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. Ce n'était pas chose aisée : la problématique que le député Masséglia a souhaité traiter est complexe. Il nous fallait apporter une solution au secteur de la presse face à ses difficultés économiques, tout en maintenant sa responsabilité environnementale sur le principe pollueur-payeur. Ce texte prévoit donc un maintien de la fusion des filières REP emballages et papier. Je crois que nous pouvons nous en féliciter tant cela apparaît comme la meilleure voie possible. Nous prenons nos responsabilités, car nous anticipons les difficultés que connaît déjà la filière papier, et nous lui permettons d'avoir un cadre qui lui apporte plus d'assise et de visibilité économique. Ainsi, nous espérons tous que la performance environnementale de la filière soit à la hauteur des ambitions. Elle le sera, car cette fusion permettra aussi d'avoir une stratégie d'écoconception commune entre des déchets qui sont déjà traités dans les mêmes centres de tri, puis recyclés ensemble. Pour la presse, l'équation était complexe, et deux solutions s'offraient à nous : la première était de construire un modèle de responsabilité propre au secteur de la presse en la sortant de la filière REP, mais tout en exigeant d'elle une contribution en nature aux contours bien définis tant sur le bénéfice et l'implication des collectivités que sur les critères environnementaux ; la seconde était de conserver la presse dans la filière REP en lui permettant de réduire sa contribution financière le mécanisme d'écomodulation conditionné à des critères de performance environnementale. Je crois sincèrement que le débat parlementaire était nécessaire sur le sujet ; les deux chambres nous l'ont prouvé. L'Assemblée nationale avait choisi la première option tout en consolidant la place et les contreparties pour les collectivités. Des amendements de différents groupes politiques avaient d'ailleurs enrichi le texte. Le Sénat, lui, a eu une autre lecture du texte, en privilégiant la seconde option. La commission mixte paritaire a finalement retenu cette seconde option et a complété la version du Sénat. Ces ajouts étaient les bienvenus, car ils viennent renforcer les garanties de progrès écologiques de la version du Sénat. Je pense notamment au fait de prévoir que les encarts donnant lieu à un bonus ne soient pas à visée promotionnelle pour le bénéficiaire, de manière directe ou indirecte. au fait de ne pas permettre de bonus si la mise à disposition d'encarts gratuits vient augmenter les quantités déchets, notamment le suremballage. C'était l'un des travers identifiés. Il n'était pas concevable de laisser un dispositif aller à l'encontre de l'ensemble des politiques publiques construites ces dernières années avec vous et qui font figure d'exemples sur la scène européenne et internationale. Je veux vous remercier, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, d'avoir mené ce dialogue constructif. Il y a quelque chose que nous sommes nombreux à partager dans cette enceinte. Nous avons tous une ambition environnementale élevée, notamment en matière d'économie circulaire. L'ambition du Gouvernement est aussi grande. Nous lançons avec ambition et fermeté les filières REP dans de nombreux secteurs. Nous avançons sérieusement sur la construction et la future mise en place d'un affichage environnemental. Nous avons réformé la filière REP textile pour la rendre encore plus performante. Nous avons fait un bond significatif dans notre performance de recyclage des emballages plastiques, notamment grâce à la généralisation du bac jaune depuis le 1 janvier 2023. Les chantiers sont encore nombreux, et ma volonté reste intacte,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues- trois semaines après l'examen en séance publique de la présente proposition de loi, nous débattons une nouvelle fois de la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et du papier, ainsi que du maintien de la presse dans ce dispositif. Absence d'étude d'impact, économie d'une deuxième lecture : nous regrettons autant de précipitation, pour une loi qui sera, quoi qu'il en soit, rétroactive. Malgré l'accord trouvé en commission mixte paritaire, je ne suis toujours convaincu ni de la simplification apportée par cette fusion ni de la solidité juridique et politique d'un texte qui mutualise les écocontributions entre producteurs de déchets. paritaire, à savoir le compromis adopté par le Sénat, maintient en vigueur ce que le droit européen nous reproche : le caractère non financier des contributions versées dans une filière REP. Je me rangerai à l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a évoqué la possibilité que le texte « donne lieu à des décisions de justice du fait de la zone d'ombre dans laquelle nous nous sommes placés ». La proposition de loi manque de clarté, et ses effets sont complexes à anticiper, que ce soit pour la presse, qui n'est pas complètement assurée d'être exonérée du caractère non financier de l'écocontribution, ou pour les autres producteurs, qui devront compenser les coûts d'une gestion des déchets dont ils ne sont pas responsables. Que devient alors le principe pollueur-payeur ? Dès lors, je regrette la suppression du rapport demandé par notre collègue Daniel Gremillet visant à évaluer l'impact de la prime accordée à la presse sur les autres contributeurs de la filière REP. De surcroît, les enjeux ne sont pas identiques pour les deux filières fusionnées. Avant de combattre la production de papier issu de la presse, luttons contre la pollution des emballages ménagers, à commencer par le suremballage en plastique. Ne nous trompons pas de combat combat ! L'argument relatif à la régression environnementale résultant d'une sortie de la REP ne nous semble pas fondé, puisque les mêmes critères de performance environnementale pouvaient s'appliquer en dehors de la REP. a d'ailleurs supprimé la précision selon laquelle ces critères ne pourront pas être moins exigeants que ceux qui existaient avant la réforme. Qu'il faille améliorer la performance du taux de collecte et de recyclage du papier, soit mais cela ne doit pas passer forcément par la réintégration de la presse dans une filière REP. Nous sommes conscients que les collectivités locales craignent un manque à gagner d'une écocontribution sur la presse qu'elles ne perçoivent pas aujourd'hui. Mais cela n'apportera pas grand-chose rapportée au coût total du service public de gestion des déchets une goutte d'eau de 15 millions d'euros à 20 millions d'euros dans un vaste océan de plus de 8,8 milliards d'euros. Certes, quelqu'un paiera : dans le premier cas, le contribuable local, dont le nombre est plus important ; dans le second cas, le lecteur, qui devient une espèce en voie de disparition. Cela se fera au profit d'une profusion de l'information rapide en ligne et des chaînes télévisées en continu, qui ne permettent pas d'aller au fond des sujets ou de s'intéresser au fonctionnement des institutions, et donc à l'exercice de la démocratie. Non, les journaux ne sont pas des déchets. Ce sont des supports culturels, comme cela a été souligné par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ; cela ne pouvait pas être la commission de la culture du Sénat, puisqu'il n'y a pas eu d'avis Le journal est tout aussi « vertueux » que le livre, et j'aurais souhaité que la commission de la culture du Sénat se prononce résolument en ce sens. Cela a été dit à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle : le maintien de la presse dans la REP visait à ne pas créer un « dangereux précédent Espérons précisément que ce texte n'en crée pas un pour intégrer ultérieurement les livres. Certaines associations demandent d'ailleurs à rompre avec la logique de l'exemption des livres et calculent qu'une écocontribution pourrait rapporter 10 millions d'euros Soyons tout de même vigilants quant au message que nous envoyons. Enfin, il a été acté à la dernière minute que le taux de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets par les éco-organismes serait renvoyé au décret. Il s'agit d'un recul supplémentaire. Mes chers collègues, je ne conteste absolument pas le bien-fondé de la REP. C'est un système qui a fait ses preuves. Je m'interroge simplement sur l'efficacité du dispositif retenu par la proposition de loi par rapport à tous les inconvénients que je viens de citer.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier. La commission mixte paritaire est parvenue à établir un texte équilibré et ambitieux pour l'économie circulaire, qui conserve de nombreux dispositifs du Sénat. Je m'en réjouis et tiens à saluer ici le travail de mes collègues, plus particulièrement de notre rapporteure, Marta de Cidrac. La proposition répond à présent pleinement aux deux objectifs qu'elle s'était fixés : d'une part, fusionner deux filières à responsabilité élargie des producteurs, celle des emballages ménagers et celle des papiers ; d'autre part, permettre, notamment pour les éditeurs de publications de presse, de moduler les contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets. Bien qu'assez technique, comme de trop nombreux textes, elle aura des effets très positifs pour le secteur de la presse et pour nos territoires. Je le disais au début de cette intervention, l'un des grands apports de ce texte est le maintien de la presse dans la filière REP. C'est un acquis décisif auquel le Sénat était très attaché, l'État ayant manqué d'anticipation en la matière. Notre collègue Didier Mandelli avait d'ailleurs souligné qu'exclure la presse de la REP aurait constitué un dangereux précédent, un manque à gagner pour le service public de gestion des déchets et une régression environnementale et juridique. Je ne peux qu'abonder en ce sens. Ensuite, si l'on entre plus au coeur des dispositions de cette proposition de loi, on peut se féliciter de la création d'un dispositif qui va bénéficier à toutes les publications de presse et aider ce secteur confronté à de graves difficultés. En effet, l'article 1 permet, des écomodulations, que le montant de la contribution financière des produits assujettis à la nouvelle REP fusionnée puisse être modulé sous forme de prime, lorsque ces produits contribuent à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets. Le bénéfice de cette modulation est ainsi conditionné au fait que les dispositifs ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages. Il est aussi précisé qu'ils ne pourront pas avoir de visée publicitaire ou promotionnelle. Les critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement pourront continuer à s'appliquer aux produits assujettis à la filière REP d'emballages ménagers et de papier. Par ailleurs, le financement et le fonctionnement du service public de gestion des déchets, géré par les collectivités territoriales, sont garantis par le texte. C'est une bonne chose au moment où les marges de manoeuvre financières de nos territoires se réduisent. Ne l'oublions des déchets reste un enjeu majeur qui soulève de nombreuses interrogations dans les territoires. Il reviendra néanmoins au pouvoir réglementaire de déterminer les taux de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers. Enfin, l'article 2 entérine l'entrée en vigueur le 1 janvier 2023 de l'article 1 et, à la suite d'un amendement de notre rapporteure, précise que les agréments des éco-organismes concernés devront être mis à jour au plus tard le 1 janvier 2024, date avant laquelle leur renouvellement est prévu. L'article 2 , issu quant à lui d'un amendement de notre collègue Daniel Gremillet, garantit un suivi effectif des impacts de la loi, en particulier celui de la modulation des contributions financières contributions financières de la filière REP pour la presse, par le biais d'un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement. Ainsi, la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier comporte de nombreuses avancées dont nous pouvons réellement nous réjouir. Elle vient répondre aux attentes des différentes filières concernées, en préservant l'intégrité de la filière REP et en y maintenant la presse. Elle n'aggrave pas les finances du service public de gestion des déchets et offre de véritables garanties environnementales. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi. La parole

Le mot sobriété, que nous entendons régulièrement, s'applique particulièrement à cette nouvelle forme de production et de consommation. Nous consommons mieux- c'est du moins ce que nous souhaitons -et, surtout, nous innovons, afin de faire évoluer nos modes de vie. L'industrie verte s'invite dans nos débats. Nos réflexions se tournent vers la décarbonation et une pollution limitée. L'économie circulaire fait partie intégrante de notre futur et de la vision d'une écologie libérale qui allie responsabilité, économie, investissements, développement et et préservation de notre environnement. Je salue le travail fourni par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, en particulier par la rapporteure de ce texte, Marta de Cidrac. Les deux assemblées sont parvenues à un accord en commission mixte paritaire, gardant beaucoup de ce que le Sénat avait inséré et renonçant à beaucoup de ce qu'il avait supprimé. La fusion des deux filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier est la bienvenue. Cela suit, de manière logique, ce que nous avions déjà organisé au moment de la loi Agec. Le point qui a particulièrement attiré mon attention est celui du sort de la presse écrite. Nous avons tous été alertés, notamment par notre presse quotidienne et hebdomadaire régionale. Leur contribution financière s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Chacun sait la situation de crise que traverse cette presse écrite, notamment régionale. Il y a la crise du papier, comme matière première, avec des prix qui augmentent significativement. En tout cas, ils augmentent assez pour que cela soit un enjeu pour le secteur. Il y a aussi un abandon du format papier en faveur du format électronique. La numérisation a également provoqué l'arrivée des réseaux sociaux dans la vie des Français. Les citoyens s'informent différemment, sur des formats qui évoluent bien plus vite que nos politiques publiques. une fois de plus alerter sur l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux. À l'heure où nous évoquons la place que prend l'intelligence artificielle dans nos vies, nous sommes inévitablement bien plus exposés aux fausses informations et aux enjeux de vérification.

Un citoyen bien informé est un électeur qui peut prendre en compte tous les paramètres d'une élection et arriver prêt devant un bulletin de vote. Voter en conscience, c'est avoir la maîtrise de notre avenir. Une presse écrite et de qualité est au fondement de notre système et de notre destin.

et mettent en lumière leur dynamisme et leur rythme de vie. Bien que le secteur soit en difficulté- nous le savons tous -, il reste essentiel. C'est dans cette perspective que le groupe Les Indépendants - République et Territoires avait été très attentif à la rédaction retenue de l'article 1 de cette proposition de loi. Nous connaissons aussi le poids, notamment financier, pour les collectivités territoriales chargées de la gestion des déchets. des déchets. L'équilibre est complexe à trouver. La rédaction finale, qui permet la modulation des contributions financières, conserve la possibilité de mise à disposition gratuite d'encarts d'information,

assuré par les collectivités et l'équilibre économique de la presse écrite, qui souffre depuis plusieurs années. Il est indispensable que les producteurs intègrent un coût de prévention et de gestion des déchets dans leur produit, pour les inciter à l'écoconception. Il s'agit de faire payer les producteurs pour les déchets qu'ils créent et de les pousser à concevoir des produits triables, recyclables ou réemployables. C'est chose faite, puisque la commission mixte paritaire a, pour l'essentiel, conservé la rédaction proposée par le Sénat. tour de passe-passe de notre rapporteure, qui maintient la presse dans la filière REP. Cette solution évite une régression environnementale, ainsi que la création d'un précédent risqué qui aurait affaibli les REP. Une telle mesure évite également- c'est peut-être l'essentiel -un manque à gagner bien lourd pour les collectivités territoriales. Elles ont besoin de ces contributions pour assurer leur service public de gestion des déchets. Ce compromis nous satisfait donc partiellement, dans la mesure où la ligne rouge n'est pas franchie : en maintenant la filière presse dans la REP papier, le principe pollueur-payeur, qui nous est cher, est préservé. Nous serons maintenant vigilants sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution en nature et veillerons à son efficacité, car la crainte d'une contagion est légitime. D'autres filières, notamment celle des emballages, pourraient prétendre à l'écomodulation. Nous espérons donc, madame la rapporteure, qu'aucune ambiguïté ne subsistera et que l'application de ce texte évitera tout risque de contagion. Nous soutenons la précision apportée en commission mixte paritaire pour que les dispositifs d'information d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets ne puissent pas avoir de visée publicitaire ou promotionnelle. Nous regrettons en revanche la suppression de la précision selon laquelle les critères qui conditionnent l'octroi de la modulation à la presse ne pourront être moins exigeants au niveau environnemental que ceux qui existaient dans le droit antérieur. Cette disposition, que les deux groupes écologistes de l'Assemblée nationale est considérée comme étant source de confusion par le député auteur de la proposition de loi. Nous pensons au contraire qu'elle levait toute ambiguïté et apportait de la clarté sur le niveau d'exigence environnementale requis. paritaire n'en est pas restée là. Elle modifie de façon substantielle un mécanisme central du fonctionnement des filières REP et des contributions des éco-organismes tels qu'ils sont prévus par la directive déchets de 2018 et par la loi Agec, à savoir la question du taux de couverture. La loi garantit le taux de couverture par la REP des coûts de gestion des déchets supportés par les collectivités : 50 % pour les papiers, 80 % pour les emballages. Or, à ce jour, ce taux n'est pas respecté par les éco-organismes : autour de 20 % pour les papiers et 50 % pour les emballages. Pour 2023, les pouvoirs publics ont évalué à environ 105 millions d'euros la somme que devrait verser Citeo aux collectivités pour couvrir 50 % des coûts des déchets papier. En 2021, cette filière a généré seulement 63 millions d'euros. fait tout de même un écart. Tout l'enjeu est donc de faire progresser d'une quarantaine de millions d'euros les versements aux collectivités. La presse exonérée représentant 17 % du gisement contribue naturellement à entretenir ce retard. La commission mixte paritaire a donc décidé de renvoyer par voie réglementaire le niveau de prise en charge des coûts des coûts de collecte et de gestion des déchets de papiers graphiques. Ils ne seront donc plus inscrits dans la loi. En d'autres termes, en renvoyant le sujet à un décret, on ouvre la voie à des négociations entre acteurs sur la répartition de la contribution globale : une facture de l'ordre de 950 millions d'euros au total pour l'ensemble de la nouvelle REP.

Quels metteurs en marché accepteront de compenser l'exonération accordée à la presse ? Comment les producteurs d'emballages combleront-ils le manque ? Est-ce juridiquement assez solide ? Nous espérons en tout cas que les collectivités ne seront pas affectées et que les coûts qui seront estimés nécessaires à la bonne gestion des déchets d'emballage et de papier ne seront pas réévalués à leur détriment. L'État doit mieux jouer son rôle de régulateur et s'assurer que les producteurs versent ce qu'ils doivent aux collectivités. Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, nous optons

du mois de février 2020 prévoyait déjà que, pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Elle prévoyait également une transition vers un dispositif harmonisé, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Désormais en place sur la quasi-totalité du territoire, ce prérequis nécessaire à la fusion des deux filières est rempli ; la fusion est désormais naturelle. Le sujet qui a le plus créé de difficultés est bien évidemment l'exemption de la presse des obligations de la filière REP ainsi fusionnée. Initialement, notre collègue député Denis Masséglia proposait d'exclure les publications de presse de la filière REP dès lors qu'elles auraient conclu une convention de partenariat, convention qu'il se proposait de créer pour tenir compte des évolutions du secteur de la presse écrite. Une telle convention conclue entre le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles professionnelles d'entreprises de presse représentatives devait préciser les modalités de mise à disposition d'espaces de communication destinés à informer le public sur la transition écologique, et ce à titre gracieux. Étaient donc dispensées du principe pollueur-payeur les publications de presse ayant signé une convention de partenariat avec l'État. Notre rapporteure a proposé une modification radicale de cette mesure avec la réintégration de la presse dans la filière REP et l'instauration d'une écomodulation pour les pour les produits de la REP contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale. En séance publique, notre groupe avait soutenu un amendement de notre collègue

Tout d'abord, la version votée pouvait contrevenir à la directive européenne relative aux déchets de 2018, entraînant un risque important de contentieux juridique. En cas de recours, la presse aurait pu se retrouver à devoir payer une écocontribution de façon rétroactive sans solution de remplacement. Ensuite, le choix des critères pouvait ouvrir le bénéfice du dispositif à d'autres organismes que celui de la presse ; c'était un précédent au sein de la REP nouvellement constituée. Ce risque d'appel d'air aurait eu des conséquences sur le montant global des écocontributions et sur les objectifs environnementaux. il imposait aux autres opérateurs d'être solidaires du secteur, alors que certains d'entre eux sont également soumis à des contraintes économiques importantes. le texte de la commission mixte paritaire confirme le maintien de la presse dans la filière REP issue de la fusion et comporte quelques modifications importantes. Il indique que les encarts d'information d'intérêt général du public ne doivent pas conduire à augmenter la quantité d'emballage ou de papier graphique et ne peuvent pas avoir de visée publicitaire ou promotionnelle. Il précise en outre que les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, l'incorporation de matières recyclées et l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Le dispositif final n'est sans doute pas parfait, mais il est néanmoins équilibré et semble, à nos yeux, acceptable pour tous. C'est pourquoi, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu durant la commission mixte paritaire et des évolutions du dispositif final aboutissant à un compromis équilibré,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de cette proposition de loi, dont l'objet initial était d'exempter le secteur de la presse de ses obligations environnementales. Alors que les filières REP créées par la loi Agec se constituent encore, notre groupe estimait que l'introduction d'une dérogation de ce type pouvait concourir à une déstabilisation du principe pollueur-payeur, auquel nous restons très attachés. Il ne s'agit pas d'opposer, d'un côté, la presse, dont nous comprenons les difficultés, de l'autre, les collectivités territoriales chargées de la gestion du service public des déchets. Le législateur a le devoir de veiller à l'application de la loi, si dure soit-elle, mais c'est la loi Ainsi, les discussions entre nos deux assemblées ont permis de maintenir le secteur de la presse dans une filière REP, ce qui est une bonne chose. Cela correspond au souhait que nous avions exprimé lors de l'examen le consensus trouvé en commission mixte paritaire est de nature à apaiser les tensions, en renvoyant finalement à l'État, par le biais de décrets, la responsabilité du niveau de prise en charge des coûts ou encore les modalités de mise à disposition d'encarts d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets. Il s'agit donc de poursuivre un régime dérogatoire qui devait s'arrêter cette année et ainsi permettre à la presse écrite de faire face à ses difficultés dans de meilleures conditions. Nous pouvons tout de même saluer le fait que la voix du Sénat ait été entendue dans le texte final. Toutefois, ce texte ne présente pas, selon nous, toutes les garanties d'un bon compromis, car il crée un précédent qui attirera mécaniquement de nouvelles demandes d'exemption émanant de secteurs fragiles au sein d'autres REP, voire d'acteurs issus de la REP papier comme l'industrie papetière, qui traverse également une importante crise tout en continuant malgré tout à payer son écocontribution. Ce n'est pas anodin, mes chers collègues, et les observateurs avertis ne s'y trompent pas, lorsqu'ils distinguent au travers de cette proposition de loi une petite révolution par la remise en cause implicite de la prise en charge des coûts du service public de gestion des déchets. Le pouvoir réglementaire aura donc toute latitude pour moduler cette prise en charge sans l'aval du Parlement. Cette modification, en dépit des précautions prises, occasionnera sans nul doute une contagion des requêtes d'exception. Dans tous les cas, il est crucial que les collectivités territoriales chargées du service public de la gestion des déchets soient étroitement associées à l'élaboration des décrets prévus par cette loi. Malgré le travail d'orfèvrerie légistique des deux rapporteurs, nous demeurons circonspects quant au texte final qui nous est soumis. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons, avec néanmoins toute la bienveillance que nous devons à Mme la rapporteure. Alors que bon nombre de filières REP se constituent parfois dans la douleur, j'espère sincèrement que cette loi ne donnera pas lieu à d'autres initiatives conjoncturelles mettant à mal le principe pollueur-payeur, qui fait consensus sur l'ensemble des travées de notre hémicycle. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi sur la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier

Certaines dispositions pour faciliter le tri sont d'ailleurs déjà lancées à la suite de l'adoption de cette loi. D'autres tardent un peu à s'étendre, comme les restrictions sur les prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres.

Les alertes sur la pollution de l'eau sont montées d'un cran ces dernières semaines. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, puisque, au-delà des pesticides que le Gouvernement laisse toujours se répandre dans nos sols et dans notre eau, les microplastiques sont aussi présents dans les cours d'eau et les océans depuis de nombreuses années. Cela nous rappelle que nos efforts sont très insuffisants et qu'il nous faut agir davantage. La fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes doit bientôt arriver. arriver. Enfin ! Cela devrait avoir un effet positif sur notre santé, avec au moins un milliard d'emballages plastiques par an évités, d'après la ministre chargée de l'écologie de l'époque.

en constatant la réduction des moyens disponibles pour assurer le recyclage et le traitement des emballages ménagers et du papier et en proposant une fusion qui devrait garantir tout à la fois une meilleure lisibilité et une réduction des coûts de fonctionnement. Permettez-moi de dire que tout n'est pas à jeter dans cette proposition de loi sur les déchets ! Cela paraît cependant un peu léger, y compris pour garantir le ramassage et le traitement des emballages et du papier, alors que les collectivités manquent la collecte finit parfois par reposer sur les usagers, qui entassent leurs déchets ou qui voient apparaître de nouveau de véritables décharges sauvages dont personne ne veut.

classique et qui favorisait les contributions en nature et pédagogiques plutôt qu'une écocontribution financière n'a pas été conservée. Une vraie réforme est à mener sur la presse écrite, comme sur la presse numérique et audiovisuelle d'ailleurs, à la fois pour favoriser l'indépendance des médias, quel que soit leur format, et pour garantir un financement nécessaire à l'existence du pluralisme de l'information et du débat public. La discussion ne peut pas porter uniquement sur la question de l'écocontribution, qui, en l'espèce, vient simplement déstabiliser un peu plus la situation économique de la presse écrite, dont nous connaissons les difficultés. C'est pourquoi le groupe CRCE s'abstiendra sur cette proposition de loi. La parole

le cadre du projet de loi de finances. La commission mixte paritaire à laquelle j'ai participé le jeudi 30 mars dernier a abouti à un accord. Sous des aspects techniques, dont le titre porte bien témoignage, le propos de ce texte était en réalité fort simple fallait-il imposer à la presse, confrontée à une hausse massive des coûts et à la crise de son modèle économique, une charge financière supplémentaire d'une vingtaine de millions d'euros de compensation de l'écocontribution en nature à Citeo à compter du 1 janvier 2023 ? d'information que j'ai présenté devant la commission de la culture au mois de juillet dernier a conclu par la négative. La presse aux abois est trop importante pour notre démocratie. Ne fragilisons pas davantage ses fondements économiques Si elle peut et doit contribuer à la révolution écologique, d'autres moyens existent. Ce constat, il faut le dire, a fait l'unanimité, à tel point que l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui reprenait et mettait en oeuvre nos recommandations. le texte de nos collègues députés reportait la charge sur les collectivités locales ; tel n'était évidemment pas notre objectif. J'avais d'ailleurs insisté dans mon rapport d'information sur la dette accumulée par l'État envers la presse, en promesses de crédits d'impôt bien mal tenues- 150 millions d'euros -et en amende à l'encontre de Google- 500 millions d'euros -, intégralement captée par le budget général.

La solution qu'elle a proposée permet de répartir la charge sur l'ensemble de la filière, ce qui me paraît plus judicieux. La presse continuera à contribuer, comme elle souhaite d'ailleurs le faire, sous forme d'encarts de sensibilisation au tri. La solution proposée, je le sais, apparaît comme moins satisfaisante pour le secteur de la presse. J'ai bien entendu les différents points de vue exprimés. Je le dis cependant clairement il y avait un fort risque que le texte de l'Assemblée nationale ne soit pas adopté du tout, un nouveau vote en dernière lecture étant pour le moins incertain. Il faut en finir avec les politiques d'autant plus généreuses qu'elles sont prélevées dans les poches des autres Dès lors, la balle est maintenant dans le camp du Gouvernement, qui devra faire en sorte que la claire volonté du législateur, exprimée par la proposition du Sénat en juillet, les votes convergents des deux assemblées et le succès de la commission mixte paritaire, soit bien respectée. La contribution de la presse, telle qu'elle sera arrêtée dans le décret prévu à l'article 1, doit se limiter à une participation en nature. J'insiste sur ce point, madame la secrétaire d'État, et j'attends de vous un engagement ferme, à même de rassurer l'ensemble de la filière.

Le scrutin est ouvert.

avancée dans sa dimension tant humaine, morale et matérielle que structurelle. L'avocat guyanais M Patrick Lingibé, actuel vice-président de la conférence des bâtonniers, dénonce « l'état parfois comateux » de la justice en outre-mer. en matière de géopolitique et de puissance maritime, sont éloignés de la République en termes de développement économique et social, mais aussi en ce qui concerne l'institution judiciaire. En 2023, les territoires d'outre-mer présentent encore de nombreuses caractéristiques d'un retard en matière démographique, sociale et économique qui, d'une part, les distingue significativement de l'Hexagone, d'autre part, pèse sur l'activité des juridictions et des services déconcentrés de l'État. L'accès au droit y est L'accès au droit y est particulièrement précaire dans un contexte de grande pauvreté et de fracture numérique, largement supérieures à ce qui est observé sur le territoire hexagonal. Le récent rapport de la Défenseure des droits le confirme clairement. L'accès au droit est un principe fondateur de l'État de droit, dont l'une des dimensions fondamentales est de garantir à tous un accès égal à l'ensemble des prestations de justice qui existent dans une société démocratique. L'aide juridictionnelle permet à celles et ceux qui n'en ont pas les moyens de faire valoir de manière effective leurs droits auprès des juridictions. Pourtant, la réalité est parfois tout autre pour les justiciables ultramarins : ils n'ont pas accès à leurs droits,

Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, des personnes placées en garde à vue n'ont aucune possibilité d'avoir un avocat à leurs côtés à cause de l'éloignement. Quant à la fracture numérique, elle existe bel et bien en outre-mer. Or le Gouvernement a annoncé un plan de transformation numérique avec un horizon fixé un ministère de la justice entièrement numérisé, donc zéro papier ... Cet objectif optimiste contraste radicalement avec les réalités ultramarines et cette digitalisation de l'institution judiciaire, pensée par la Chancellerie, est aujourd'hui profondément inadaptée pour les outre-mer. Un rapport

chronique des moyens dévolus à la justice en outre-mer a fait l'objet de nombreuses alertes et préconisations. Je prends l'exemple de la revalorisation de l'unité de valeur au profit des avocats ultramarins, qui doivent parfois se déplacer en avion ou en bateau pour aller défendre Une telle mesure permettrait d'apporter une réponse à des justiciables qui se trouvent privés d'avocats en l'absence de tout dispositif de prise en charge. Dans un contexte de défiance importante vis-à-vis des institutions, les services judiciaires sont, en raison de leur mission régalienne, particulièrement exposés aux tensions sociales et à l'insécurité chronique que connaissent certains territoires ultramarins. La crise de confiance est majeure dans l'Hexagone ; elle est totalement désastreuse en outre-mer. Le dernier épisode dans le scandale du chlordécone- un non-lieu décidé après dix-sept années de procédure -va assurément augmenter cette crise de confiance envers la République et sa justice. L'argumentation juridique n'a malheureusement

et étendue, pour la première fois, aux outre-mer que 58 % des Ultramarins affirment qu'il est difficile de faire valoir ses droits. La situation des établissements pénitentiaires y est particulièrement préoccupante. En 2019, à deux reprises, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié en urgence des recommandations, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, à la suite de la constatation de violations graves des droits fondamentaux des personnes incarcérées dans les centres pénitentiaires de Rémire-Montjoly, en Guyane, et de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nous savons que les prisons françaises sont surpeuplées, mais

soit une densité carcérale de 123 %, légèrement supérieure à celle de l'Hexagone, qui est de 119,7 %, avec 56 219 places disponibles pour 67 299 détenus. Mais la problématique carcérale ultramarine ne réside pas dans son taux de suroccupation que dans les conditions indignes et inhumaines de détention, qui ont souvent été décriées. D'ailleurs, il est à relever que, dans l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 janvier 2020 2020 condamnant la France pour des traitements dégradants et de mauvaises conditions de détention, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,

La prise de poste y est parfois extrêmement difficile, surtout pour les magistrats et les greffiers sortant directement des écoles de formation. De façon générale, les services publics ultramarins posent des problèmes

des agents affectés dans ces territoires doivent être prises en compte de façon systématique pour faciliter la prise de poste., un mécanisme d'avance sur rémunération et un accompagnement individualisé pour l'installation sur place sont indispensables. Le taux d'absentéisme dans les services judiciaires atteint un niveau supérieur à la moyenne nationale, le taux de rotation est particulièrement élevé et l'ancienneté moyenne est bien inférieure à celle que l'on constate à l'échelle nationale.

aux populations des différents territoires d'outre-mer. Monsieur le ministre, votre gouvernement est-il prêt à répondre aux problématiques qui se posent de façon régulière dans nos territoires ? La parole

Je précise d'emblée que je ne pourrai pas, comme vous le savez, répondre sur les affaires en cours, pas plus que n'aurait pu le faire le garde des sceaux. Mais c'est avec plaisir que je vais tenter d'apporter des éclairages sur vos préoccupations. Comme dans d'autres domaines, l'action du Gouvernement en la matière est empreinte à la fois de volontarisme et de pragmatisme. Il nous faut regarder les actions d'aujourd'hui et non pas seulement les rapports publiés voilà plusieurs années

La politique de conciliation est essentielle, je vous rejoins sur ce point. Dans chacun des deux départements antillais, deux conciliateurs ont pu être recrutés en 2022. Cela est encore insuffisant, je le conçois, mais les juridictions poursuivent des campagnes de recrutement. Les Antilles bénéficieront, comme l'ensemble du territoire, du large déploiement de la politique de l'amiable, l'une des suites des États généraux de la justice. Nos concitoyens souhaitent que leurs litiges puissent avancer. Or, parfois, la médiation ou d'autres modes de règlement des différends répondent mieux à leurs préoccupations que le recours à la justice en tant que telle.

68 personnels contractuels sont arrivés en outre-mer dans le cadre du déploiement de cette justice de proximité. La Chancellerie a bien pris en considération les recommandations du Défenseur des droits et procédera prochainement à un recensement des audiences foraines existantes et des besoins concrets des juridictions en la matière.

Au-delà, ce sujet rejoint celui du coût de la vie dans les outre-mer, sujet qui, comme vous le savez, fait lui aussi l'objet de perspectives précises que le ministre de l'intérieur et des outre-mer C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la revalorisation de l'unité de valeur ne fait pas partie des évolutions envisagées. Je souhaite plus largement revenir sur l'intitulé du débat de ce jour : l'état de la justice Mon collègue garde des sceaux est pleinement conscient que cet état n'est pas toujours parfait, pas plus qu'il ne l'est d'ailleurs dans l'Hexagone, mais cela résulte, vous le savez bien, d'une très longue histoire. Les hausses importantes du budget de la justice au cours des dernières années permettent cependant d'entrevoir de potentielles améliorations. De nombreuses créations de postes ont eu lieu : 108 postes de magistrats et de fonctionnaires ont été créés dans les services judiciaires depuis 2018, dont 71 dans les deux dans l'administration pénitentiaire, on est passé entre 2020 et 2023 de 2 800 à 2 932 postes en outre-mer, soit autant de postes supplémentaires permettant aux Ultramarins, très nombreux dans l'administration pénitentiaire, de revenir exercer leurs fonctions sur le territoire dont ils sont originaires.

Ainsi, l'aide à l'installation est permise pour les magistrats et greffiers depuis l'an dernier, par le biais d'un marché public. Un contrat de mobilité est aussi possible pour des postes de magistrat souffrant d'une absence de candidats : pour ces postes, le passage outre-mer est un véritable tremplin pour la carrière, avec l'assurance après trois ans de revenir dans l'Hexagone sur l'un des cinq postes sollicités en partant. Avant les choix de postes, une formation intitulée existe pour sensibiliser ceux qui sont intéressés. Des pôles spécialisés existent désormais à la direction des services judiciaires, pour sensibiliser aux spécificités de ces territoires. Des interventions sur les postes outre-mer sont désormais systématiques au moment des choix des postes, à la sortie de l'École nationale de la magistrature ou de l'École nationale des greffes. Le ministère de la justice a donc désormais parfaitement compris que, pour que la justice outre-mer fonctionne, il faut que les personnes venant y contribuer soient conscientes des spécificités du territoire dans lequel elles arrivent, et qu'elles soient accueillies, accompagnées et formées. Le ministère de la justice contribue également à l'emploi outre-mer. Ainsi, je veux ici mettre en lumière que 28 % des surveillants recrutés depuis 2017 sur l'ensemble du territoire national sont originaires des territoires ultramarins : c'est un chiffre important. un concours national d'affectation locale est en cours pour recruter sept greffiers à Mayotte et dix en Guyane. De même, les outre-mer sont largement concernés par le plan de 15 000 places de prison, visant à moderniser

Parvenir à l'égalité réelle des droits et des services pour tous nos concitoyens, où qu'ils résident, impose des obligations. L'accès de tous à une justice de qualité en fait partie. ministre, souhaiterais-je vous interroger sur l'aide juridictionnelle, qui n'est pas suffisamment adaptée à la réalité des territoires ultramarins. C'est un point que le Parlement connaît bien, car les difficultés liées à l'aide juridictionnelle reviennent chaque année à l'occasion de l'examen de la loi de finances. finances. Mon collègue Stéphane Artano s'inquiète en particulier du problème des frais de déplacement des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Leur défraiement n'est prévu que pour la Polynésie française.

Je souhaite donc attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'ajuster les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle notamment que cette indemnisation soit relevée dans tous les territoires où l'accès aux juridictions est particulièrement difficile. Monsieur le ministre, doit-on rappeler que l'égalité est au coeur de notre pacte républicain ?

Saint-Barthélemy fait face à une nette augmentation de la délinquance. Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ont connu une hausse de 50 % entre 2021 et 2022, les portant à 123 faits. Les escroqueries ont, quant à elles, connu une hausse de 25 %, de même que les atteintes aux biens. Pour autant, malgré une convention

pour faire face à ce phénomène relativement nouveau par son ampleur. Les effectifs judiciaires ont ainsi progressé moins vite que les besoins. La première des préoccupations porte sur le rajeunissement des prévenus.

dans la zone. Une part importante des délits est liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiants. En la matière, la rapidité de la sanction judiciaire contribue à l'indispensable message de fermeté en matière de sécurité, sur une île comme Saint-Barthélemy. Depuis trois ans, les contentieux civils sont également en forte hausse. Saint-Barthélemy concentre 70 70 % des contentieux des îles du Nord. Ceux-ci portent principalement sur des baux d'habitation, des demandes d'expertise ou des successions. Monsieur le ministre, ma question est donc simple : une mise à niveau des effectifs est-elle envisagée à court terme pour Saint-Barthélemy ? La parole est à M. le ministre

On y retrouve néanmoins des problématiques similaires. L'état de la justice dans les outre-mer laisse en effet apparaître une surpopulation carcérale parfois plus importante que dans l'Hexagone, mais également une insécurité extrêmement préoccupante dans certaines collectivités. De nombreuses juridictions souffrent d'un manque d'attractivité. Il est bien difficile, dans ces conditions, d'assurer le remplacement des magistrats mutés. Alors que les déserts médicaux, économiques et démographiques côtoient parfois des déserts judiciaires, la question de l'accès au droit se pose pour beaucoup de nos compatriotes ultramarins. Les difficultés géographiques et démographiques sont nombreuses. Chaque territoire tente de les résoudre le mieux possible. Ainsi, en Polynésie française, une dotation existe, afin de prendre en charge les frais de déplacement des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En revanche, à Wallis-et-Futuna, les accusés sont bien souvent défendus devant les cours d'assises par des citoyens défenseurs qui ne sont pas des avocats. En effet, l'aide juridictionnelle ne couvre pas aujourd'hui l'ensemble des frais de déplacement des avocats venant de Nouméa. Monsieur le ministre, quelles solutions peuvent être envisagées pour permettre à tous nos concitoyens d'être assistés ou représentés par un avocat chaque fois que cela est nécessaire ? Serait-il possible d'étendre le dispositif polynésien à l'ensemble des territoires ultramarins ? Il est indispensable de garantir à chaque enfant de la République

ressorti des États généraux de la justice, qui se sont tenus l'an dernier, était attendu, même si leurs conclusions sur l'état de la justice dans notre pays n'ont pas surpris grand monde : 70 % des Français estiment que la justice n'a pas les moyens suffisants pour faire son travail. La justice est malade ; c'est en effet le résultat d'une très longue histoire.

dématérialisation à outrance, l'apport d'assistants de justice- postes non pérennes -, l'envoi pour des périodes limitées de magistrats en renfort dans ces juridictions en souffrance ou encore la construction de places de prison comme marqueurs chiffrés d'une justice qui reprend vie soient la réponse appropriée. Dernièrement, le vice-président de la Conférence des bâtonniers a pu s'exprimer sur le sujet, relevant la faible place octroyée aux outre-mer dans le rapport issu des États généraux de la justice. Il préconise, pour parfaire la connaissance du territoire,

La spécificité démographique, géographique et sociologique de ces territoires riches de plus de 2,7 millions d'habitants doit être mieux prise en compte. Aussi ma question portera-t-elle sur l'assistance des personnes placées en garde à vue, dont on sait que certaines n'ont parfois, pour des raisons d'éloignement, pas la possibilité d'avoir un avocat à leurs côtés. Le Gouvernement compte-t-il réfléchir à la mise en place de dispositifs sécurisés d'assistance en garde à vue lorsque les distances rendent la venue d'un avocat impossible dans des délais raisonnables ?

Monsieur le ministre,

dans le rapport issu des États généraux de la justice. C'est peu lorsque l'on sait que les terribles constats qu'il dresse sont plus graves encore dans ces territoires. Entre particularismes géographiques, pauvreté, fracture numérique, barrières linguistiques, défaut d'attractivité et insécurité, les outre-mer cumulent les difficultés. En outre, l'accès à la justice y est complexifié d'effectivité de certains droits essentiels, comme l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ou l'indemnisation des frais de déplacement des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin ou encore Saint-Laurent-du-Maroni

est démontrée depuis leur création. L'inspection générale de la justice (IGJ) soulignait néanmoins, en octobre 2020, la nécessité de bâtir un plan stratégique d'actions à la fois communes et propres à chaque territoire ultramarin. que l'outre-mer compte 13 territoires répondant à 4 catégories juridiques différentes, avec, pour chacun d'entre eux, un cadre institutionnel différent ! Cela suppose, selon l'IGJ, de développer une fonction prospective jusqu'à présent peu investie par l'administration centrale. quelles suites le Gouvernement entend-il donner à cette recommandation pour injecter, désormais, les sucres lents dont nous avons tant besoin ?

de la Contrôleure sur le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, en Guyane, dont je vous lirai seulement les titres : « La surpopulation est chronique », « Les conditions d'hébergement sont indignes

se traduira par le déploiement de 400 gendarmes mobiles supplémentaires et la venue de la CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, pour effectuer des reconduites à la frontière. est effectué entre l'immigration et la délinquance et l'instrumentalisation dont fait l'objet l'institution judiciaire, mise au service d'une politique pénale décidée par le ministère de l'intérieur, ne sont pas acceptables.

Nos magistrats du siège doivent demeurer indépendants et se tenir loin d'une politique pénale expéditive et du tout-répressif. Des reconductions aux frontières expéditives, je dirai même systématiques, se font forcément

Où sommes-nous ? Il nous faut réagir ! Les opérations de reconduites à la frontière et de destruction des habitats indignes qui sont engagées et se poursuivront sont naturellement conduites, croyez-le, dans le strict respect du droit des personnes mineures.

les instances administratives et judiciaires locales entretiennent au quotidien des relations très fluides avec les avocats mahorais et réunionnais dans le cadre du traitement du contentieux lié aux opérations de déconstruction et de reconduite. Tous les services de l'État sont mobilisés pour faire face à la situation sécuritaire et migratoire, en agissant en priorité contre les délinquants, les réseaux criminels et les passeurs, et pour offrir des conditions d'accueil dignes aux ayants droit. Nous faisons tout pour respecter le droit judiciaire. La priorité est de faire juger rapidement les personnes interpellées,

dans les outre-mer, « l'accès au droit est particulièrement précaire dans un contexte de pauvreté et de fracture numérique largement supérieures à ce qui est observé sur le territoire européen de la France ». En effet, en raison de l'état des infrastructures de réseau et d'un taux d'illectronisme plus élevé, comme l'a souligné Victoire Jasmin, les Ultramarins n'ont pas accès aux services numériques dans les mêmes conditions que dans l'Hexagone. Nos collègues de la délégation aux outre-mer Stéphane Artano, Viviane Artigalas et Nassimah Dindar en faisaient déjà le constat dans un rapport d'information déposé le 9 juillet 2020, qui a montré les effets dévastateurs de la fracture numérique en période de confinement dans certaines parties, exclues et isolées, Or, lors de sa présentation du plan d'action pour la justice le 5 janvier 2023, le garde des sceaux a fixé « un horizon clair pour 2027 : un ministère de la justice entièrement numérisé », avec un « objectif zéro papier ». Ce but optimiste contraste radicalement

de ces territoires un accès numérique effectif à la justice et au droit ? La parole

et mes collègues Alain Marc et Thani Mohamed Soilihi, seize recommandations, dont le renforcement des moyens humains du tribunal judiciaire, la création d'une véritable cour d'appel et la construction de locaux adéquats. Le garde des sceaux s'est rendu à Mayotte en mars 2022 pour y faire une série d'annonces qui vont en partie dans le sens du rapport sénatorial. Mais, alors qu'un jeune greffier a dénoncé ses conditions de travail dans une lettre avant de tenter de mettre fin à ses jours, les recrutements d'agents qui ont été annoncés pour répondre aux besoins sont certes louables, mais insuffisants. Il faut augmenter, d'une part, les moyens du parquet, d'autre part, les moyens d'instruction des juridictions mahoraises. Plus encore, de la création d'une véritable cour d'appel en lieu et place d'une simple chambre détachée l'on nous oppose régulièrement le fait que l'organisation actuelle semble satisfaisante au regard du faible volume des affaires traitées, c'est là faire fi de la réalité mahoraise.

Face aux nombreux problèmes liés au caractère archipélagique de la Guadeloupe, des mesures spécifiques doivent être envisagées par le Gouvernement pour revoir et adapter les modalités d'indemnisation des frais inhérents à l'exercice des fonctions des conseillers prud'homaux de notre archipel.

condamnées. La parole est à M. Gérard Poadja. Monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen par le Sénat du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, j'avais appelé l'attention du Gouvernement sur le fait que nous étions le seul territoire de la République à ne pas disposer disposer sur notre sol d'un centre d'accès au droit. La loi du 22 décembre 2021 a réparé cette injustice en prévoyant la création d'un centre d'accès au droit en Nouvelle-Calédonie à destination des personnes les plus éloignées.

Néanmoins, l'état du bâti demeure très vétuste et sous-dimensionné. Monsieur le ministre, ce constat pose évidemment la question du respect de la dignité des détenus, quand ceux-ci sont entassés, parfois à cinq ou six, dans une cellule de douze mètres carrés. À ce jour, l'État a été condamné par la justice administrative à verser plus de 700 000 euros d'indemnités. Par ailleurs, à la suite des rapports de Mme la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, les magistrats de l'ordre judiciaire ont prononcé des remises en liberté au motif que ces conditions de détention constituaient un traitement dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

tenue. La parole est à M. Bernard Jomier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France a été condamnée à de multiples reprises ces dernières années, aussi bien par sa propre justice que par la CEDH, pour les conditions indignes de détention qu'elle impose dans ses prisons, y compris en outre-mer. Mes collègues Jean-Pierre Sueur et Pierre Frogier l'ont souligné. L'état de ces prisons n'est que l'un des symptômes du mal qui frappe la justice dans son ensemble dans les outre-mer. Une enquête, réalisée en 2021 pour le Conseil national des barreaux, révélait que 58 % des Ultramarins- jusqu'à 70 % en Guyane -considèrent qu'il leur est difficile de faire valoir leurs droits, ce qui constitue une proportion deux fois plus élevée qu'en métropole. Cette injustice résulte d'une multitude d'inégalités. Comment ne pas s'alarmer, par exemple, de l'absence pure et simple d'avocats dans certaines situations, en raison d'un manque d'accompagnement de l'État pour les aider dans leurs déplacements ?

la part du financement des services publics dans notre pays représentait 18,1 % du PIB en 1980, contre 18 % aujourd'hui, alors que la population a très nettement augmenté. L'intégralité de la hausse de la dépense publique a profité aux transferts vers les entreprises. Dans le même temps, la population des outre-mer est passée de 1,4 million à 2,7 millions d'habitants. Le gouvernement auquel vous appartenez refuse de revenir sur la moindre des nombreuses exonérations fiscales et sociales

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le tribunal de Saint-Martin est un tribunal de proximité. Sa juridiction couvre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il dépend du tribunal judiciaire de Basse-Terre, notamment en termes de moyens et de ressources humaines. Ce tribunal dispose des plus importantes dérogations de la République.

survient avec beaucoup de retard en raison du sous-effectif du greffe. La solution, urgente et nécessaire, serait d'accorder au tribunal de proximité de Saint-Martin son autonomie totale de tribunal judiciaire et les moyens qui vont avec. En effet, monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi qu'il revient à l'État d'assumer la continuité territoriale et l'égalité devant la justice. Il n'est pas normal que les Saint-Martinois ne bénéficient pas, comme tous les Français de l'Hexagone, d'un accès effectif à la justice de leur pays. Seriez-vous prêt, monsieur le ministre, à pallier ces difficultés par des réformes législatives ou réglementaires

un pouvoir central unique, une structure administrative homogène et l'uniformité du droit applicable sur l'ensemble de notre territoire. Notre Constitution est donc potentiellement rétive à la reconnaissance des particularismes juridiques. Toutefois, ce principe d'indivisibilité n'a pas empêché- et c'est heureux ! -l'existence d'une République plurielle. Si cette pluralité implique une certaine plasticité de nos institutions, elle ne doit pas conduire à renier nos principes. Avant tout, je tenais à rappeler

N'oublions pas que les outre-mer ont une histoire particulière et que le rapport à l'État français n'a pas toujours été simple dans l'ensemble de ces territoires qui composent notre République. L'expression étatique, notamment par le biais de ce

Nous réagissons trop fréquemment selon un biais hexagonal, reconnaissons-le. Dès lors, l'adaptation de nos dispositifs n'est pas toujours optimale. Par ailleurs, le comité des États généraux de la justice indique que les caractéristiques démographiques et socio-économiques des outre-mer les distinguent significativement de la métropole.

de l'Hexagone. Toutes celles et tous ceux qui connaissent ici l'outre-mer, même sans y habiter, savent ces difficultés et ce qu'elles représentent sur le plan de la délinquance. Toutes ces inégalités doivent être prises en compte, ainsi que les spécificités liées à l'éloignement de ces territoires et à leurs particularités géographiques. Il n'est pas possible de se dire, en 2023, que les justiciables n'ont pas tous et toutes les mêmes droits et les mêmes accès au droit. Nous nous réclamons de l'État de droit. Or la justice est la clé de voûte de ce système. L'État, seul, est à même d'exercer cette fonction, afin d'en garantir l'impartialité.